La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du vendredi 7 juin 2019 a été publié sur le site internet

réunie ce jour a décidé, en accord avec le Gouvernement, de modifier l'ordre du jour des mercredi 12, jeudi 13 et mardi 18 juin. Le mercredi 12 juin, à quinze heures, aura lieu la lecture devant le Sénat de la déclaration de politique générale du Gouvernement. En conséquence, l'espace réservé au groupe communiste républicain citoyen et écologiste,

qui sera suivie d'un débat et d'un vote par scrutin public à la tribune. En conséquence, l'examen de la proposition de résolution visant à clarifier et actualiser le règlement du Sénat est reporté au mardi 18 juin, à quatorze heures trente. Y a-t-il des observations ?

alinéa 4, du règlement, tout ou partie d'un texte peut être renvoyé, sur décision du Sénat, à la commission, pour une seconde délibération, à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée par le Gouvernement. Le Gouvernement accepte-t-il cette demande de seconde délibération ?

sur la question de l'interruption volontaire de grossesse, ou IVG, je ne peux être suspectée d'aucune façon. Chacun le sait, je suis particulièrement attachée à l'amélioration des droits sexuels et reproductifs des femmes. Le délai de recours à l'IVG n'est pas le même entre les pays, mais les systèmes de prise en charge des IVG ne sont pas toujours organisés comme le nôtre. L'objectif premier est que toutes celles qui le souhaitent doivent pouvoir bénéficier d'une IVG sûre et de qualité, quelles que soient leurs conditions et dans tous les territoires. Je serai intraitable et me battrai inlassablement, parce que les menaces sont constantes- l'actualité internationale nous l'enseigne tous les jours. Nous devons ainsi poursuivre nos efforts pour assurer une offre diversifiée de proximité réelle et accessible de façon permanente, répondant aux besoins des territoires en matière d'IVG. J'aurai l'occasion de revenir devant les parlementaires pour présenter les résultats de l'enquête lancée auprès des agences régionales de santé pour identifier les difficultés d'accès éventuellement rencontrées. C'est pour cela que j'ai soutenu l'amendement de Mme la sénatrice Laurence Rossignol rétablissant le rapport du Gouvernement au Parlement sur l'accès à l'IVG. Ce rapport sera rendu en fin d'année. J'estime à présent en conscience et en responsabilité que les conditions dans lesquelles le Sénat s'est prononcé vendredi dernier pour allonger le délai pour recourir à une IVG n'étaient pas satisfaisantes. Elles n'étaient pas satisfaisantes compte tenu des circonstances particulières du vote. Elles n'étaient pas satisfaisantes, parce que le projet de loi est centré sur l'organisation des soins. Je sais que cette demande d'allongement du délai d'IVG est soutenue par le planning familial, acteur incontournable du droit des femmes, et j'en recevrai les membres pour discuter avec eux de l'accès à l'IVG. En acceptant la seconde délibération demandée par la commission des affaires sociales, je veux réunir les conditions ... Lesquelles ? ... pour que ce débat légitime ait lieu dans le bon cadre et en assurant l'ensemble des échanges que l'importance du sujet exige. Cela ne peut pas être traité dans ce projet de loi et dans les conditions dans lesquelles le débat s'est déroulé. Très bien ! Pour cette raison et sans préjudice du débat et des justes questions posées sur l'accès effectif à l'IVG, débat qui devra se tenir dans un cadre plus adapté,

seconde délibération. Je salue les applaudissements soutenus dont Mme la ministre vient de bénéficier de la part de la droite, sur un sujet aussi sensible et aussi clivant entre la droite et la gauche que l'est celui de l'IVG.

Le scrutin est ouvert.

décidé. Conformément à l'article 43, alinéa 5, de notre règlement, délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter un nouveau rapport La commission va donc se réunir pour présenter un rapport. J'interroge la commission sur la durée de la suspension qu'elle estime nécessaire

ne se rattache au projet de loi que de manière très ténue, du fait de la présence, à l'article 17 du texte déposé à l'Assemblée nationale, d'une mesure de simplification prévoyant la suppression de l'obligation pour les professionnels de santé concernés de réaliser, à des fins statistiques, un bulletin papier pour chaque interruption volontaire de grossesse. Il intervient sans qu'aucune concertation préalable ait été menée sur ce sujet, notamment avec la communauté scientifique et médicale. Ce n'est pas dans ces conditions ni dans ces circonstances, au terme de l'examen d'un texte portant

émane non pas de quelques sénatrices ou de quelques sénateurs, mais de professionnels de la santé ou de structures, comme le planning familial, qui accompagnent les femmes ayant recours à une IVG.

sont enceintes et que leur retard de règles est le signe d'une grossesse, et non un déséquilibre de leur contraception. Enfin, les mineures, les jeunes filles, elles, ne savent même pas ce qui leur arrive et n'osent pas en parler. Voilà de bonnes raisons d'allonger de deux semaines le délai d'IVG, comme cela se pratique dans bien d'autres pays.

Votre liste aux élections européennes a promu le « pacte Simone Veil », le « bouquet législatif », la solidarité entre les femmes de tous les pays d'Europe pour les meilleures lois sur l'IVG. Quel message envoyez-vous

sur un sujet aussi important et sensible, la première des choses à faire est, me semble-t-il, de prendre de la hauteur et d'agir de façon dépassionnée. Je rappelle tout d'abord que le droit à l'IVG a été considérablement amélioré ces dernières années. En 2001, les délais pour pratiquer une IVG ont été portés de dix à douze semaines. En 2013, l'IVG est devenue gratuite pour toutes les femmes. En 2014, la notion de détresse a disparu. En 2016, le délai minimal de réflexion d'une semaine a été supprimé, les sages-femmes pouvant désormais pratiquer des IVG médicamenteuses et les centres de santé des IVG instrumentales.

C'est pourquoi nous n'avons pas participé non plus au vote sur la seconde délibération. En effet, comme nous l'a expliqué Mme la ministre, le Sénat a rétabli l'article 27, qui prévoit la remise d'un rapport sur l'accès effectif à l'IVG et sur les difficultés d'accès à l'IVG dans les territoires, y compris les refus de certains praticiens praticiens de pratiquer une IVG. Sur la forme, il nous paraît indispensable de prendre le temps d'une réflexion très approfondie sur un tel sujet, notamment, mes chers collègues, au regard de ce qui se pratique chez nos voisins. Il y a mieux, il y a pire. Le présent texte ne nous semble donc pas constituer le bon véhicule législatif.

Ce débat sur le prolongement du délai de l'IVG doit ainsi relancer les interrogations sur les circonstances et les facteurs qui conduisent plus de 200 000 femmes par an à vouloir interrompre leur grossesse. Le CCNE considère que le débat éthique se situe en amont et pas seulement dans l'allongement du délai prévu par la loi. » La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, j'interviendrai non pas en tant que sénateur, mais en tant que praticien, radiologue, J'ai aidé beaucoup de femmes ayant pour projet d'interrompre une grossesse. J'étais à côté d'elles, j'ai ressenti leur douleur. À douze semaines, c'est un embryon qui mesure 6,5 centimètres de distance crânio-caudale où l'on ne voit que le bourgeon germinal. À quatorze semaines, nous sommes face à un foetus, dont on a 99 % de chances de dépister le sexe.

tous, je souhaite que nous ayons un véritable débat sur ce sujet de fond. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pour ma part, je ne prendrai pas part au vote.

fondamental, au détour de n'importe quelle loi : nous ne les laisserons jamais le brocarder

des experts, dont le planning familial fait partie, mais aussi dans le cadre du débat parlementaire, qui, je dois dire, nous honore. La preuve en est que, au sein du groupe LaREM, nous ne partageons pas tous le même point de vue, comme

Je pense que vous rendez un très mauvais service aux Français, aux Françaises et la France. Vous vous rangez dans le camp des grands conservateurs du vaste mouvement conservateur qui se développe partout en Europe,

La réalité, c'est que les Anglais, les Espagnols, les Islandais ne sont pas moins humanistes, moins soucieux de la vie humaine, moins respectueux de la vie en général que nous, Français.

Vous accroissez les inégalités, mais, au fond, c'est la philosophie même de ce grand mouvement d'émancipation que vous remettez en cause, avec, comme d'habitude, les mêmes arguments, les mêmes votes qu'à l'époque, et ce peu de temps après la panthéonisation

C'est totalement caricatural, et je refuse absolument d'être classée dans la catégorie des conservateurs qui voudraient revenir sur le droit de l'IVG. C'est un sujet de fond qui mérite un débat serein, digne et respectueux des uns et des autres, qui ne saurait être traité au détour d'un amendement présenté un vendredi matin.

que, parce que nous ne sommes pas d'accord, parce que nous cherchons à comprendre, nous ne serions que d'horribles conservateurs

Le délai d'IVG allongé par le Sénat : " un vrai plus " pour les femmes ». J'en extrairai les mots suivants : « Cet amendement pourrait bien changer la vie de nombreuses femmes. Quand on découvre qu'on est enceinte et qu'on prend la décision d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse (IVG), il faut garder en tête les délais. Jusqu'à maintenant, l'IVG chirurgicale n'était possible que jusqu'à la douzième semaine de grossesse il fallait se lancer dans les démarches sans vraiment traîner et trouver l'établissement adéquat. C'est parfois beaucoup plus compliqué qu'auparavant, puisque, depuis de nombreuses années, certains établissements publics ou privés qui pratiquaient l'IVG ont fermé. Et les délais d'attente se révèlent souvent trop longs. Certaines femmes n'ont parfois d'autres choix que de se rendre à l'étranger pour avorter, mais toutes ne peuvent se le permettre côté financier. C'est pour cela

La loi Veil a été votée après vingt-six heures de débat. Ce n'est pas au détour d'un amendement que l'on peut tout changer. Je pense qu'un grand texte, madame la ministre, honorera le Parlement.

Monsieur Karoutchi, votre intervention a clarifié quelques points, mais je me demande comment nous, parlementaires, allons pouvoir justifier l'annulation du vote de vendredi auprès

la vie de ces femmes et nous permet de préserver un droit à l'intervention volontaire de grossesse dans de bonnes conditions. La parole

C'est le cas en France depuis la révision du délai par la loi du 4 juillet 2001, mais également en Allemagne, en Belgique, en Italie, au Danemark, en Autriche. Les quelques pays qui autorisent l'avortement au-delà de ce délai ne le font qu'à des conditions très restrictives. Au Royaume-Uni, en Espagne ou en Finlande, l'avortement doit en effet être justifié par des raisons socioéconomiques, autrement dit un viol,

Si le délai de douze semaines à compter du début de la grossesse a été retenu par la plupart des pays européens, c'est également, évidemment, pour des raisons de faisabilité technique. Le geste médical nécessaire pour une IVG après ce délai n'est plus le même et le protocole doit être révisé compte tenu des risques importants pour la femme enceinte après ce délai. Plus qu'une question de délai, c'est donc bien un problème d'accès

lorsqu'il s'agit d'orienter ou de rediriger les patientes, en leur rappelant qu'ils doivent sensibiliser très tôt les patientes sur le respect des délais pour procéder à l'IVG, en tenant compte du délai pour manifester son consentement. Il faut aussi renforcer la formation à l'IVG, par exemple en permettant à plus de médecins généralistes de suivre un diplôme interuniversitaire de gynécologie ou un DU en orthogénie, ce qui implique de soutenir plus d'initiatives en ce sens, comme au travers du réseau entre la ville et l'hôpital pour l'orthogénie en Île-de-France. en outre d'établir une cartographie précise des structures pratiquant l'IVG. Enfin, il faut sanctionner les professionnels de santé qui, après avoir exercé leur clause de conscience, méconnaissent l'obligation qui leur est faite de réorienter les patientes vers un médecin ou un centre susceptible de pratiquer une IVG. La commission avait souhaité inscrire un pouvoir de pénalité pour les organismes d'assurance maladie à l'encontre des professionnels ne respectant pas cette obligation, mais le groupe CRCE s'y était, à l'époque, refusé. Je

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est clos. J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement

Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues,

La séance est reprise. En votre nom à tous, mes chers collègues, je tiens à saluer la mémoire des sauveteurs de la Société nationale de sauvetage en mer, la SNSM, qui ont perdu la vie vendredi dernier au large des Sables-d'Olonne et ont porté jusqu'au sacrifice ultime l'honneur, le dévouement et le courage. Ils s'appelaient Yann Chagnolleau, Alain Guibert et Dimitri Moulic. Au nom du Sénat tout entier, nous avons une pensée pour eux, pour la famille des disparus, mais aussi pour les sauveteurs dont la vie a été épargnée.

Merci,

Les circonstances du drame sont désormais connues : la mer était totalement démontée. Pourtant, lorsqu'ils ont reçu le signal de détresse relayé par le Cross Étel,

parce que c'est leur raison d'être- et même de mourir, malheureusement. Depuis que cette terre est battue par la marée sans fin de la vie et de la mort, tous ceux qui portent secours pour sauver des vies savent qu'un jour ils peuvent mourir. Mais rien n'a plus d'importance que leur devoir, accompli parfois jusqu'à l'ultime sacrifice. Le Président de la République a décidé

qui sait reconnaître les héros. Vous êtes ému par le sens du devoir et par le courage dont font preuve des concitoyens qui n'en attendent rien, si ce n'est le sentiment d'accomplir une mission pour laquelle ils s'engagent.

un département où l'on sait que la mer donne beaucoup et reprend parfois. Tous les gens de mer, tous ceux qui ont grandi près de la mer, tous ceux qui l'aiment savent que rien n'est plus fort que les éléments.

Union Centriste. Ma question s'adresse à M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire. Une émotion vive et sincère s'est emparée de la ville des Sables-d'Olonne, de la Vendée et de l'ensemble de la communauté maritime. Le vendredi 7 juin, alors que la tempête Miguel fait rage, sept marins expérimentés, sauveteurs bénévoles de la station SNSM des Sables-d'Olonne, ont fait naufrage à bord du canot tout temps. Animés par la solidarité des gens de mer, ils allaient porter assistance à un bateau de pêche. Des murs d'eau ont eu raison du canot qui s'est retourné, une première fois, une deuxième et une troisième, fatale. Trois hommes sont morts. Quatre hommes parviendront à rejoindre la côte dans des conditions invraisemblables. Hier, 15 000 personnes leur ont rendu un hommage poignant à travers une marche silencieuse. Ces hommes et ces femmes s'engagent bénévolement pour sauver des vies. Ils méritent notre respect. Ils sont sauveteurs en mer, pompiers, membres de la protection civile et remplissent des missions de service public. Le canot était le bateau de réserve de la station. Cette embarcation de 1986 est sortie dans des conditions de mer dantesques. canot n° 1, pour sa part, est en réparation depuis de nombreux mois, parce que l'association SNSM, composée de 8 000 bénévoles, subventionnée à 80 % par des dons, n'a pas les moyens de renouveler tout son matériel navigant. Monsieur le ministre, j'en appelle à une nécessaire et urgente prise de conscience collective afin de doter ces hommes et ces femmes qui s'engagent pour les autres de moyens financiers et matériels suffisants, pour que soit préservé et consolidé le statut de bénévole et qu'un accompagnement des familles des victimes soit assuré. Je vous prie

Madame la ministre, cette situation ne surprend personne. Si les moyens alloués depuis quelques années ont augmenté sensiblement, le recours des patients aux services d'urgences a augmenté davantage Bien souvent, il s'agit plus de consultations non programmées que de véritables urgences, notamment en périodes d'épidémie de grippe. Mais il est vrai aussi que, pour bon nombre de Français, le service des urgences est parfois le seul recours possible. La suppression de la permanence des soins en ambulatoire en 2003 n'a sans doute rien arrangé, mais l'on sait qu'il est toujours difficile de revenir en arrière. Et si le personnel des urgences est au bord du burn-out, les médecins de ville ne sont pas mieux lotis, avec 50 à 60 heures de travail hebdomadaires, hors permanence des soins.

Personnellement, je ne crois pas à l'efficacité de la mesure d'un forfait de réorientation, car il faudrait déjà une préconsultation pour affirmer le caractère non urgent de l'acte à effectuer. De surcroît, cela constituerait un manque à gagner pour les urgences. Je rappelle que le coût moyen de l'acte d'admission pour l'assurance maladie est de 150 euros, quelle que soit la gravité. Le Sénat n'a d'ailleurs pas voté cette mesure. Ayons l'humilité d'admettre que nul ne possède la solution miracle, surtout- disons-le clairement -à moyens constants. Certes, les mesures que vous proposez- maisons médicales de soins non programmées et hôpitaux de proximité -apporteront des solutions à moyen et long terme, madame la ministre. Mais, à court terme, que pouvez-vous proposer ?

la souffrance des personnels dans les urgences est une réalité. Les difficultés de travail sont anciennes, mais elles se sont aggravées. Le constat est clair

J'ai ajouté 300 millions d'euros non utilisés en 2018, que j'ai réalloués aux hôpitaux en mars 2019. J'ai également augmenté pour la première fois depuis dix ans les tarifs hospitaliers, non pas ce que les gens payent, mais ce que la sécurité sociale rembourse aux hôpitaux pour leur activité. Je montre ainsi aux personnels que je suis à leurs côtés, en attendant la réorganisation du système de santé, objet de la loi qui va être soumise à votre vote tout

et à éviter de trop longues attentes aux urgences, en permettant à des professionnels paramédicaux de prescrire, par exemple, des actes de radiologie ou de biologie. Enfin, j'ai demandé aux agences régionales de santé d'allouer des moyens supplémentaires

Les lignes d'aménagement du territoire ne représentent que 0,3 % du trafic des aéroports de Paris, mais elles sont vitales pour certains départements enclavés, difficilement accessibles par le rail ou la route. Afin de compenser le déficit de ces lignes aériennes, à côté de la puissance publique, les collectivités les financent de façon très importante, au maximum de leurs possibilités. Il va sans dire que la hausse des taxes sur le kérosène, kérosène, tout à fait légitime en raison du réchauffement climatique qui nous touche de plein fouet, accroîtrait encore le déficit de ces lignes et risquerait de les mettre en danger. On parle beaucoup de différenciation dans les politiques publiques territoriales. C'est d'ailleurs l'une des dispositions prévues par le projet de loi de réforme constitutionnelle. Dans cette logique, le kérosène utilisé pour le fonctionnement de ces lignes ne pourrait-il pas être détaxé, afin de permettre à nos territoires isolés de maintenir leur activité économique et de se développer ? À défaut, l'État ne pourrait-il pas prendre à sa charge le surcoût financier d'une mesure extrêmement préjudiciable pour nos territoires déjà fragilisés ? Le rôle de l'État est de protéger les plus faibles afin de ne pas aggraver une fracture territoriale que ne supportent plus nos concitoyens.

Depuis trois mois, les services d'urgence sont engagés dans un mouvement de grève pour alerter la population et le Gouvernement sur les conditions intolérables d'accueil et de prises en charge des patients. Selon le collectif Inter-Urgences, 95 services d'urgences sont actuellement en grève pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail, un manque de moyens, mais surtout la dégradation des soins offerts aux patients. Ce mouvement de grève est une mobilisation d'intérêt général au service de la dignité humaine. Madame la ministre, vous avez annoncé la création d'un soutien financier aux établissements confrontés à un surcroît d'activité et à des afflux exceptionnels, mais les services d'urgences sont confrontés à cette situation toute l'année. Qu'allez-vous faire si le service d'urgences du centre hospitalier de Lens ferme ses portes cet été, comme le craignent les personnels ? Allez-vous faire appel au service de santé des armées, comme l'a évoqué le président de la Fédération hospitalière de France ? Qu'allez-vous faire, madame la ministre, face à l'urgence sociale et sanitaire de nos hôpitaux ? La parole

l'ensemble des professions de santé qui vont être impactées par ces difficultés particulières pour préparer la permanence des soins.

Vous m'interpellez par ailleurs plus généralement sur les difficultés des urgences. Je l'ai dit, ces services sont aujourd'hui le symptôme d'un système de santé qui dysfonctionne à la fois en amont,

à faciliter l'accès à des soins de ville non programmés. C'est l'engagement que prendront notamment les professionnels de santé qui intégreront une communauté professionnelle territoriale de santé.

90 services d'urgence sont en grève. Les personnels sont dévoués, compétents, mais fatigués, usés et souvent au bord des larmes quand les admissions croissent chaque année, jusqu'à atteindre 21 millions selon les tout cela sans augmentation de moyens, au contraire. Près de 50 % des médecins exerçant aux urgences sont contractuels, donc précaires. Pourtant, les signaux d'alarme n'ont pas manqué. Le décès de Micheline à Lariboisière après 14 heures sur un brancard n'était pas le moindre

d'euros. À qui la faute ? Madame la ministre, en dehors des 700 millions d'euros que vous leur attribuez, pris sur les gels de l'an passé, quels moyens efficaces entendez-vous mettre en oeuvre pour ouvrir un horizon plus souriant aux personnels hospitaliers et aux Français qui, majoritairement, soutiennent leur mouvement ?

La réforme que je propose est financée. Je viens de dégager plus de 700 millions d'euros pour l'hôpital, avec une augmentation des tarifs pour 2019. J'ai demandé en outre qu'une partie de ce budget

plastronniez lorsque le budget était en équilibre grâce aux efforts de la gauche pendant des années. Maintenant qu'il est en équilibre, vous puisez à pleines mains dans les caisses de la sécurité sociale et vous n'avez plus de moyens pour satisfaire les besoins de l'hôpital

qui s'appliquent à plus d'une trentaine de pays, à des personnes morales et physiques, à des marchandises ou à des moyens de transport. Les pays concernés voient leur économie affectée par ces mesures. Mais ces sanctions pèsent lourdement sur les entreprises françaises travaillant à l'international. Le transport maritime, en particulier, est lourdement touché. L'environnement commercial devient de plus en plus instable et complexe pour les opérateurs économiques, en raison de la multiplication des cibles. Les sanctions évoluent très vite, si vite même qu'un bateau en pleine mer peut se trouver immobilisé du jour au lendemain, avec des conséquences financières considérables. L'armateur doit alors se séparer de la cargaison, mais aussi du navire, pour éviter des sanctions à son encontre et à l'encontre de ses partenaires, banquiers ou assureurs. Au quotidien, nos entreprises doivent s'assurer que leurs opérations ne sont pas visées par de nouvelles sanctions sans préavis. Elles s'imposent des règles et des procédures strictes et extrêmement lourdes. Elles consacrent des heures à remplir des questionnaires, notamment sur l'historique Ces conditions les amènent trop souvent à ne pas pouvoir honorer leurs contrats. Du fait de l'évolution rapide des régimes d'embargo et de sanction sans préavis, nos entreprises sont exposées à un risque permanent. Comment peut-on simplifier et stabiliser leur environnement ? Nos entrepreneurs se sentent pris en otage par les décisions du Trésor américain, qui se livre à une guerre commerciale qui ne dit pas son nom. Le renforcement du pouvoir des autorités de contrôle est considérable. Le cas le plus emblématique en la matière est celui des décisions de l'OFAC. Monsieur le secrétaire d'État, dans un contexte commercial instable, quelles mesures le Gouvernement compte-t-il prendre afin de mieux protéger les activités et les intérêts des armateurs et des groupes multinationaux français dont l'activité est menacée par des sanctions imprévisibles ? La

mot pour mot, je n'ai rien à retirer de votre question. Nous nous battons avec la même philosophie que la vôtre avec nos collègues européens. Très clairement, les États membres de l'Union européenne ont un rendez-vous majeur avec l'exercice de leur souveraineté économique. Il n'est pas acceptable que nos alliés nous dictent là où il est bon ou pas de commercer pour les entrepreneurs européens. De ce point de vue, un certain nombre de mesures ont été prises il y a déjà une vingtaine d'années- je pense au règlement de 1996 -pour faire en sorte que les mesures prises en application de la loi Helms-Burton par les États-Unis ne puissent pas trouver à s'appliquer. Nous devons aller plus loin encore aujourd'hui. D'ailleurs, c'est

de nos outils, notamment le règlement de 1996. Également, nous allons faire en sorte d'affirmer tout simplement cette puissance européenne. Nous n'avons pas peur de revendiquer que cet espace de 500 millions d'habitants et de consommateurs doit peser encore et toujours plus. Bastiat disait il y a un peu plus d'un siècle que, là où le commerce passe les frontières, les soldats ne la passent pas. Quelques jours après avoir commémoré dans l'unité cette belle leçon des Alliés à l'été 44, souvenons-nous que nous devons faire en sorte que le commerce international connaisse une désescalade des tensions pour ne pas menacer la stabilité tout simplement.

Elle porte sur les turbulences récentes, mais fortes, que traverse le groupe Renault. Déjà ébranlée par plusieurs mois de tensions, à la suite du départ rocambolesque de Carlos Ghosn, l'alliance est de nouveau éprouvée par la discussion, puis le retrait apparent ou réel- vous nous le direz -d'une offre de fusion faite par le groupe Fiat. La compétitivité et la conquête d'opportunités par Renault ont toujours été, au fil des différents gouvernements, une priorité industrielle et stratégique pour notre pays. Or un potentiel rapprochement pour le moins précipité avec Fiat n'aurait probablement pas atteint ces objectifs : la proposition de Fiat s'appuyait sur une valorisation au rabais de Renault, donnait les coudées franches à la famille Agnelli dans la gouvernance de la nouvelle entité fusionnée et divisait par deux la part de l'État dans l'actionnariat. Au-delà de ce « deal » enterré peut-être aussi soudainement qu'il a été envisagé, je souhaiterais que vous nous éclairiez sur les opportunités que vous pourriez encore voir à cette éventuelle alliance entre ces constructeurs assez similaires, deux constructeurs qui chassent souvent dans les mêmes zones géographiques et sur les mêmes gammes de voiture. Quels sont les risques également en matière d'emploi, de gouvernance et d'alliance ? Pouvez-vous nous indiquer si vous poursuivez, officiellement ou pas, avec le groupe Renault la discussion ? Quelles seraient vos conditions pour un accord ? Quelles garanties pourriez-vous demander ? Enfin, il n'est pas impossible que ces allers et retours avec Fiat mettent en péril l'alliance entre Renault et Nissan. La tiédeur de Nissan devrait d'ailleurs nous inviter à la prudence : le groupe japonais s'est abstenu lors du vote au sujet de la fusion. Le ministre Bruno Le Maire s'est rendu au Japon la semaine dernière à l'occasion du G20 Finances pour tenter d'apaiser les relations entre les deux groupes, et Nissan, qui tiendra le 25 juin prochain son assemblée générale, vient d'apprendre par courrier que Renault s'opposait à la nouvelle gouvernance du groupe japonais. Comment entendons-nous, nous État actionnaire, soutenir le groupe Renault pour sortir du blocage actuel et rétablir un dialogue de qualité constructif au sein de l'alliance ? La parole

actionnaire de Renault à hauteur de 15 %, l'a accueillie avec ouverture et a travaillé de manière constructive et professionnelle avec l'ensemble des parties prenantes. Je crois que c'est ce qu'on est en droit d'attendre de tout actionnaire au conseil d'administration de Renault. Nous avons été évidemment soucieux des intérêts stratégiques de l'industrie automobile française. Bruno Le Maire avait immédiatement fixé quatre conditions préalables- qui devraient de toute éternité nécessairement être réunies si d'autres dossiers de cette nature, ou différents, devaient se présenter -à l'approbation de l'opération par l'État. La première condition, c'est la réalisation de cette opération dans le cadre de l'alliance entre Renault et Nissan. Il n'y a pas d'ambiguïté : si Renault a un partenaire stratégique qui est Nissan, il convient que cette alliance soit respectée et que chacun soit à l'aise autour de la table du conseil d'administration. C'est aussi la clé de la réussite des vrais projets industriels. La préservation des emplois industriels et des sites industriels en France est la deuxième condition, les autres conditions étant une gouvernance respectueuse des équilibres de Renault et de FCA et la participation de ce futur ensemble industriel à l'initiative des batteries électriques engagée avec l'Allemagne, tant cette initiative est également primordiale pour l'avenir de l'industrie automobile européenne. Je veux dire ici que des progrès significatifs ont été faits sur les trois derniers éléments. C'est la question d'un délai additionnel pour s'assurer du soutien de l'ensemble des parties prenantes, notamment du soutien explicite de Nissan, qui a amené FCA à retirer son offre. L'État prend acte de cette décision. Je crois que nous n'avons pas à rougir d'avoir posé ces conditions, qui étaient de bon sens, de bon aloi et, je le redis, Pour la suite, Bruno Le Maire était effectivement au Japon ces derniers jours. Il faut conclure ! Il a vu son homologue japonais, M. Seko. Il peut vous garantir l'attachement de la France et du Japon à l'alliance. Ce sujet était bien à l'agenda et nous allons progresser. La parole

profondes et des origines parfois anciennes. La sociologie des « gilets jaunes » et les résultats des dernières élections européennes témoignent de cette double fracture sociale et territoriale. Le grand débat a été l'occasion pour le Président de la République et pour le Gouvernement d'avoir une écoute bienveillante et de renouer un dialogue plus direct et plus approfondi avec les élus locaux. Il a suscité chez beaucoup d'entre eux l'espoir d'être enfin compris. Le Président de la République a annoncé dès janvier et confirmé en avril un nouvel acte de décentralisation accompagné d'une révision ou d'une adaptation de la loi NOTRe et d'une déconcentration des services de l'État, et ce dans un souci de proximité, d'efficacité et, même, d'économies. fin d'avril, monsieur le Premier ministre, vous annonciez pour le mois de juin une étape de concertation sur la déconcentration des décisions prises par l'État et sur une nouvelle organisation territoriale de l'État. Mais jusqu'à présent, rien de très concret sur la décentralisation et la révision de la loi NOTRe. Pourtant, le transfert de nouveaux blocs de compétences, des assouplissements dans l'organisation des compétences entre collectivités, le rétablissement de l'intérêt communautaire ou encore la différenciation territoriale sont des sujets sur lesquels les élus locaux ont de fortes attentes de mesures concrètes. Pouvez-vous, monsieur le Premier ministre, nous indiquer, sur ce volet décentralisation et collectivités locales, le périmètre, les grandes orientations, la méthode et le calendrier envisagés par le Gouvernement pour engager cette réforme essentielle pour nos territoires ?

les derniers mois que nous avons vécus ont mis en avant à la fois les inquiétudes sociales, mais également les inquiétudes territoriales. Et à l'issue de ce grand débat national, le Président de la République s'est engagé sur deux éléments très importants : le premier, c'est consolider l'exercice des mandats locaux, en particulier le mandat de maire ; le second, c'est d'ouvrir un nouvel acte de décentralisation. Pour répondre concrètement à votre question, deux projets de loi seront présentés. S'agissant de l'engagement

de les remercier et de leur témoigner toute la considération que la République leur doit bien évidemment. Ce projet de loi sera présenté dans les prochaines semaines en conseil des ministres pour une adoption avant les élections municipales de 2020. Le Premier ministre aura l'occasion de détailler

de nos concitoyens. Pour ne prendre que cet exemple, évidemment qu'il faut plus décentraliser la politique du logement, parce que c'est lorsque vous élisez votre maire que vous vous demandez si ce dernier peut impacter celle-ci. Et lorsque vous voyez que cette politique est encore trop conduite par zonage, vous vous dites que cette décentralisation est importante. pour la réplique. Merci, monsieur le ministre. Il y a quelques mois seulement, nous avons été un peu échaudés par une loi sur l'eau et l'assainissement, avec un assouplissement en forme de report d'échéances, ce qui a laissé un goût amer au Sénat. J'espère qu'à l'avenir les positions du Gouvernement prendront mieux en compte le principe de subsidiarité tel qu'il a été défini par le Président de la République lorsqu'il déclarait en début d'année : « Je crois que l'on a besoin de remettre de la responsabilité au plus près du terrain.

vous n'êtes pas sans savoir que les services d'urgence des hôpitaux français, en proie à une crise profonde depuis de nombreuses années, sont aujourd'hui à bout de souffle. Il y a douze ans déjà, un rapport de notre Haute Assemblée les décrivait comme le « miroir grossissant des dysfonctionnements de l'ensemble de notre système de santé de santé ». Vous aviez annoncé dès votre prise de fonction prendre ce problème à bras-le-corps. Mais qu'en est-il réellement ? Force est de constater que la situation s'aggrave et s'amplifie de jour en jour face à l'inadéquation entre le nombre de passages, les moyens alloués et la disponibilité des lits d'aval. Malgré les nombreux plans déjà mis en place ou annoncés, on ne peut que constater leur inefficacité chronique. Résultat : les personnels de santé des urgences multiplient les mouvements de grève sur tout notre territoire. Peut-on les blâmer au vu des chiffres et de la dégradation de leurs conditions de travail ? Certainement pas. En vingt ans, les urgences ont vu leur fréquentation doubler. Nos personnels sont confrontés, chaque jour, à la multiplication des agressions tant verbales que physiques. Car qui dit saturation des services, dit exaspération des patients et épuisement des personnels soignants, qui se sentent délaissés. Nos professionnels de santé réclament à juste titre davantage de moyens humains et financiers. Alors, vous me répondrez certainement que la loi Santé, votée à l'Assemblée nationale et en cours de délibération au Sénat, porte la double ambition de mieux répartir l'accès aux soins et de libérer les établissements hospitaliers sous tension. Mais les mesures annoncées ne devraient voir le jour qu'en 2022 : ce sera déjà trop tard ! Il y a urgence, madame la ministre, pour nos urgences ! Nous ne pouvons plus attendre, car nous parlons ici de notre bien le plus précieux, la santé des Français, mais aussi celle de nos personnels de santé, qui n'en peuvent plus, tant physiquement que psychologiquement. Alors, ma question est simple : quelles mesures d'urgence allez-vous initier pour éviter que d'autres drames ne surviennent, pour agir enfin et pour faire face à cet enjeu majeur de santé publique qui est sous votre responsabilité ?

évidemment, vous avez raison : le système est en tension depuis de nombreuses années et l'augmentation du nombre des passages aux urgences n'a fait qu'aggraver les choses. J'ai souhaité accompagner les hôpitaux cette année avec, en particulier, un dégel de crédits, avec un refinancement de 300 millions

crédits nouveaux soient fléchés particulièrement vers des services d'urgences. En réalité, la situation est très variable d'un service à l'autre, tout comme le sont les besoins. Dans certains cas, il manque des médecins ; dans d'autres, plutôt des professionnels paramédicaux dans d'autres cas encore, les locaux sont extrêmement vétustes et trop petits pour accueillir le flux de malades. Il faut donc pouvoir donner à chaque hôpital, à chaque site, la réponse appropriée. J'ai donc demandé aux agences régionales de santé d'accompagner les hôpitaux en tension. Certains ne le sont pas : il y a beaucoup de services d'urgences en France qui fonctionnent avec moins de 15 000 passages par c'est-à-dire moins de deux passages par heure. Il faut aussi être attentif à ce que les budgets accompagnent les sites les plus en difficulté. C'est ce que nous allons faire dans les semaines qui viennent. Au-delà de la mission nationale confiée au président du Conseil national de l'urgence hospitalière, le professeur Pierre Carli, et au député Thomas Mesnier afin de repenser notre système d'urgences pour le refonder, j'annoncerai très concrètement comment cette offre d'accompagnement va aller vers les établissements et vers les professionnels, dont je ne néglige pas la charge de travail, à la fois physique- nous le savons, vous comme moi, parce que vous êtes un professionnel de santé aussi -et émotionnelle : aux urgences, il est extrêmement difficile, en effet,

socialiste et républicain. Ma question s'adresse à l'ensemble du Gouvernement. La France compte plus de 1,3 million de jeunes qui ne sont ni à l'école, ni à l'université, ni en apprentissage et ni en emploi. Concernant l'outre-mer, et particulièrement la Martinique, l'apprentissage est rendu encore plus difficile en raison du tissu économique principalement constitué de microentreprises, ce qui rend l'accueil d'apprentis très difficile et maintient les jeunes et leurs familles dans l'angoisse et le doute permanent. Pour être totalement transparent, mesdames, messieurs les ministres, je suis sollicité toutes les semaines par de jeunes Martiniquais- et leurs familles -, qui, face à l'indispensable nécessité d'une alternance, ne trouvent pas d'entreprise et sont contraints d'abandonner leurs études. D'ailleurs, si l'on prend en compte l'ensemble de l'alternance, apprentissage et professionnalisation, on observe une baisse des effectifs de 4,1 % par rapport à février 2018. La réforme de l'apprentissage voulue par le Gouvernement, qui s'accompagne de la mise en place d'un nouveau statut de l'apprenti, théoriquement plus attractif pour les jeunes, ne semble pas faire consensus localement, principalement parce que les conditions requises pour obtenir la « prépa apprentissage » sont identiques à celles de l'apprentissage lui-même- nécessité d'obtenir un contrat d'apprentissage. donc des jeunes qui n'arriveront pas à trouver de contrat de travail dans le cadre de ce nouveau dispositif ? Une enquête de Studyrama révèle ainsi que 84 % des sondés, entre le bac et bac+5, ont trouvé la recherche d'une entreprise très difficile. Je souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement en la matière pour nos jeunes ultramarins, qui se sentent totalement abandonnés.

Je vous remercie de votre question, qui met en lumière les difficultés relatives à l'emploi, à l'insertion professionnelle et, plus largement, à la formation des jeunes, en particulier dans les outre-mer, notamment en Martinique. Je partage avec vous le constat d'un chômage qui frappe plus durement non seulement les jeunes, mais également les territoires d'outre-mer par rapport au reste du pays. du pays. Cette difficulté, nous la connaissons évidemment et nous avons souhaité agir depuis le début du quinquennat pour y apporter des réponses. Vous vous en souvenez sans doute, le Livre bleu des outre-mer, en 2018, avait fléché 700 millions d'euros du programme d'investissement dans les compétences spécifiquement pour les outre-mer, apportant ainsi un soutien fort à la formation professionnelle, qui est un vecteur de reprise d'emploi. Nous avons également, en avril 2019, étendu le dispositif des emplois francs sous l'autorité de Muriel Pénicaud, d'Annick Girardin et de Julien Denormandie.

C'est la raison pour laquelle une ordonnance spécifique découlant de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel sera dédiée aux outre-mer. Cette ordonnance a fait l'objet d'une large concertation, laquelle continue aujourd'hui avec les élus locaux à la fois pour dresser un diagnostic et proposer des solutions. Elle précisera les règles de gouvernance et de déploiement dans les outre-mer des dispositifs relatifs à l'apprentissage. Je veux vous assurer, monsieur le sénateur, de notre préoccupation constante sur ce sujet et de notre volonté de développer l'apprentissage également dans les outre-mer. La parole

depuis vendredi dernier, un scandale alimentaire- un de plus -secoue notre pays : celui des steaks hachés de très mauvaise qualité distribués aux plus démunis. Cette affaire est choquante à double titre. D'abord, car elle constitue une faute morale intolérable, en visant nos concitoyens se trouvant en situation de précarité. Ensuite, parce qu'elle constitue une fraude, une tromperie sur la qualité des produits achetés. Les médias l'ont rappelé, plusieurs acteurs sont intervenus dans cette chaîne, que je qualifierai de particulièrement longue : le fonds européen d'aide aux plus démunis, qui soutient financièrement les États de l'Union l'État, qui a confié à FranceAgriMer l'organisation d'un appel d'offres ; puis, enfin, une entreprise financière retenue pour le marché, mais qui s'appuie sur une autre entreprise, polonaise cette fois-ci, pour son approvisionnement en viande. En outre, ce qui demeure regrettable, c'est que seul le prix ait été retenu comme critère dans cet appel d'offres. D'ailleurs, je m'interroge : comment se fait-il que le ratio entre le prix total d'achat et le poids de la viande vendue n'ait pas appelé l'attention des pouvoirs publics la secrétaire d'État, l'État ne devrait-il pas mieux imposer la prise en compte du critère lié à la qualité dans l'attribution de ces marchés ? au nom du bon sens écologique, économique et solidaire la DGCCRF a effectivement annoncé vendredi matin avoir découvert une tromperie sur la qualité des steaks hachés distribués par une entreprise française à des associations de soutien aux plus démunis. Je veux d'abord être nette sur deux points. C'est une affaire qui est le fait d'escrocs cyniques qui pensaient pouvoir agir en toute impunité. C'est raté,

Je veux également revenir sur les faits. D'abord, ce sont les associations qui ont été extrêmement réactives, puisque, dès qu'elles ont constaté que la marchandise ne correspondait pas au cahier des charges, elles nous l'ont signalé et en ont suspendu la distribution. Ce faisant, elles nous ont permis de

Comme les autres, il a, bien sûr, pour ambition de construire le système de santé de demain. Il s'inscrit dans le prolongement du plan Ma santé 2022, présenté par le président Macron, en septembre 2018, qu'il décline en texte de loi. Il s'agit, tout d'abord, de réformer les études médicales avec une mesure phare, qui sonne tout de même comme un effet d'annonce, je veux parler de la suppression du Comme le précise le président de la conférence des doyens de médecine, « cette suppression ne va pas changer massivement le nombre de médecins formés

Toutefois, d'autres épreuves sélectives, à préciser par décret, remplaceront cette dernière. Restent cependant des inconnues : d'abord, la capacité des universités et des hôpitaux d'accueillir les étudiants constitue un facteur limitant et pose aussi une question budgétaire pour l'État l'orientation des étudiants Parcoursup à la sortie du baccalauréat ; enfin, les besoins en professions médicales des territoires qui seront à l'origine de discussions entre universités et agences régionales de santé, À l'autre extrémité du cursus, l'examen classant national, qui sera lui aussi supprimé à la fin du deuxième cycle, est remplacé par un dispositif visant à s'assurer du niveau de connaissances des étudiants tout en prenant en compte les compétences et le parcours des candidats pour le choix de leur spécialité. Si une réforme des études médicales a pour ambition première de mieux former les étudiants, elle tend aussi à offrir aux territoires un meilleur accès aux soins. Comme vous l'avez dit vous-même, madame la ministre, cela « ne réglera pas le problème de la démographie médicale viens à mon deuxième point, le problème des déserts médicaux. Je n'aime pas cette expression tant elle recouvre des réalités fort différentes : les zones rurales, en effet désertifiées, pas seulement par leurs médecins, mais aussi par les services publics les banlieues, quant à elles surpeuplées, mais où les médecins hésitent à s'installer du fait de problèmes de sécurité ; enfin, les hôpitaux eux-mêmes où de nombreux postes ne sont pas pourvus. En fait, ce dont nous manquons, c'est moins de médecins que de temps médical. L'exercice de la médecine a changé parce que la société a changé. Disons-le clairement, ce point a été l'objet de vifs débats au Sénat, chambre des territoires. Deux opinions s'affrontent : les tenants de la coercition ou, du moins, d'une régulation musclée, et ceux de l'incitation, d'ailleurs déjà mise en place avec des résultats divers. Personnellement, je suis convaincu de l'inefficacité des mesures coercitives, en particulier du conventionnement sélectif, instauré, il est vrai, pour les professions paramédicales, mais dans le cadre d'une négociation conventionnelle.

pour objet de faire de la dernière année de troisième cycle une année de professionnalisation, de pratique ambulatoire en autonomie. Il visait à permettre, en particulier, aux étudiants en troisième année de diplôme d'études spécialisées, DES, de médecine générale d'exercer en tant que médecin adjoint. On pourrait même imaginer une quatrième année à ce DES sans que cela implique d'ajouter une année supplémentaire aux DES des autres spécialités, sauf à considérer- ce n'est pas mon cas -la médecine générale comme une non-spécialité ou une sous-spécialité. Non, par cette proposition, le Sénat ne brade pas la formation des médecins ! Il considère, au contraire, qu'une dernière année professionnalisante est une chance de consolider leur formation, tout en favorisant la construction de leur projet professionnel. Pour autant, je suis bien conscient qu'une telle mesure ne réglera pas tout, mais elle pourrait apporter une amélioration à un dispositif forcément plus global. implique, de la part des étudiants en fin de formation, ainsi que des jeunes médecins, une prise de responsabilité populationnelle en plus de la responsabilité individuelle qui est déjà la leur. C'est à ce prix que nous sauverons la médecine libérale ou ce qu'il en reste, mais le veut-on vraiment ? Faute de quoi, nous pourrions bien arriver à une médecine salariée, que beaucoup appellent déjà de leurs voeux, doublée d'une médecine déconventionnée, pour le coup redevenue vraiment libérale et qui ferait la joie des sociétés d'assurance dans leurs diversités. Ce chapitre est loin d'être clos ! Autre dispositif visant à améliorer l'offre de soins dans les territoires : les communautés professionnelles territoriales de santé qui élaboreront les projets territoriaux de santé soumis à l'ARS. Il s'agit de faire en sorte que les professionnels s'approprient ce dispositif et d'éviter qu'une grille de l'ARS ne s'applique sur les territoires. Cela implique, comme je l'ai déjà évoqué, une prise de conscience populationnelle de la part des acteurs, laquelle suppose de dégager du temps médical, non plus clinique, mais de santé publique, après des journées de travail déjà épuisantes. Quant aux hôpitaux de proximité, nous aurions certes aimé avoir plus de précisions concernant leur contenu, mais il y va du choix de légiférer par ordonnance sur ce sujet. Ils me paraissent l'outil nécessaire et efficace pour assurer une gradation des soins, ainsi qu'une meilleure interpénétration ville-hôpital-secteur médico-social. Si, comme on peut l'espérer, cet outil est rapidement mis en place, il pourrait apporter une réponse aux besoins des territoires en matière de premier niveau de soins, véritable interface entre médecine de ville et établissements de santé de recours. Encore faudra-t-il en définir le bon format, le bon plateau technique, le bon contenu en ressources humaines : urgences, actes techniques ne nécessitant pas d'anesthésie, imagerie, biologie ... Nous comptons sur vous, madame la ministre, pour répondre, dans les meilleurs délais, à ce juste questionnement. Il ne me reste pas assez de temps pour aborder dans le détail le titre III du projet de loi qui vise à développer l'ambition numérique en santé. Je rappellerai simplement les inévitables questions éthiques liées à ce big data de la santé, questions soulevées par un avis du Comité

à quatorze semaines. Rassurez-vous, je n'y reviendrai pas, j'ai déjà dit tout le mal que j'en pensais ! Mais cette seconde délibération ne grandit pas le Sénat ! Ce propos liminaire terminé, je tiens à remercier les administratrices et administrateurs

En renforçant la lutte contre les conflits d'intérêts dans la formation continue des médecins par les industriels de santé, en alignant la durée du zonage des zones sous-denses- trois ans -sur celle de l'internat de médecine générale, en annulant les règles de captage d'eau d'origine souterraine et en supprimant l'expérimentation de l'exercice libéral dans les centres de santé, les dispositions de nos amendements ont apporté des modifications positives, mais bien maigres pour contrecarrer les mesures régressives de ce projet de loi. De plus, nous déplorons que nos amendements tendant à défendre et à améliorer le droit à l'IVG- je pense à l'autorisation de la pratique de l'IVG instrumentale par les sages-femmes, ou encore à la suppression de la double clause de conscience -aient été retoqués. Je vous rappelle, mes chers collègues, que notre groupe défend la constitutionnalisation du droit à l'IVG qui est sans doute une solution pour garantir et protéger ce droit. Plus globalement,

D'ailleurs, aujourd'hui même, à l'appel de l'intersyndicale CGT, FO, SUD, CFE-CGC, les personnels sont de nouveau rassemblés devant le ministère des solidarités et de la santé pour se faire enfin entendre, et ils ont tout notre soutien Nous regrettons votre entêtement, madame la ministre, votre refus de prendre en compte la gravité de la situation, après des décennies de réduction des dépenses de personnel, de report des investissements, de fermetures de services et de suppressions de lits.

qui n'en peuvent plus. Ils vous réclament la création de 10 000 postes dans les services d'urgence, la réouverture de lits d'aval en prévision de cet été et, enfin, une revalorisation salariale de 300 euros nets par mois. Comment rester inébranlable au sujet des demandes de renfort de personnel quand on sait que les besoins se situent à hauteur de 100 000 emplois dans les hôpitaux publics et de 100 000 emplois par an, sur trois ans, dans les Ehpad ? Les primes que vous avez annoncées face à la mobilisation grandissante de toutes les catégories de personnels des urgences ne sont pas de nature à éteindre la colère

pleuvent. Mais pourquoi personne n'envoie les gendarmes chercher les directeurs d'ARS pour négocier et les directeurs réquisitionnés pour dialoguer ? Lors des débats sur les déserts médicaux, des sénatrices et des sénateurs de différents groupes politiques ont défendu des mesures de régulation de l'implantation des médecins libéraux dans les déserts médicaux. Et bien que les questions de l'attractivité de la médecine de ville et du maintien des services des hôpitaux de proximité soient liées entre elles, les mêmes parlementaires sont restés silencieux, voire n'ont pas jugé utile d'être présents dans l'hémicycle lors du vote de l'article 8 prévoyant la réforme des hôpitaux en trois niveaux, avec des hôpitaux de proximité vidés des services d'urgence, de gériatrie, de chirurgie et de maternité Seul notre groupe s'est opposé à la nouvelle architecture et à la future organisation des hôpitaux, en proposant, comme en 2014, un moratoire contre toutes ces fermetures et une autre définition de l'hôpital de proximité. Nous pensons, en effet, que le maillage d'hôpitaux de proximité doit être maintenu et développé avec des services d'urgence, fonctionnant 24 heures sur 24, de médecine, de chirurgie, d'obstétrique, de soins de suite et des structures pour les personnes âgées en lien avec la médecine de ville, le réseau de centres de santé et la psychiatrie de secteur, qui est décidément, une nouvelle fois, la grande oubliée de ce projet de loi. N'attendez pas, madame la ministre, avant de vous apercevoir que nous avions raison comme avions raison comme aujourd'hui pour la suppression du ! Nous déplorons que, avec la complicité bienveillante de la majorité sénatoriale, la philosophie de ce texte ait été confortée, à savoir affaiblir toujours davantage ce qui fait la colonne vertébrale de notre système de santé public : l'hôpital. Notre groupe s'est battu pied à pied pour une autre logique. Dans le fond, le Gouvernement répond au personnel hospitalier en grève : « soigne et tais-toi ».

Mais, visiblement, mes chers collègues, plus le Gouvernement restreint les prérogatives des législateurs que nous sommes et plus vous votez les textes qu'il présente ! Je vous invite à lire ou à relire le de La Boétie, très instructif. Vos critiques sont souvent acerbes pour poser le diagnostic d'un système de santé à bout de souffle, mais vous êtes d'accord avec les remèdes proposés, qui, de réforme en réforme, transforment le patient en client et l'hôpital en entreprise ! De cette politique-là, nous ne voulons pas ! Nous ne nous tairons pas, nous voterons contre ce projet de loi et nous continuerons à défendre, comme nous nous y sommes engagés lors de notre tour de France des hôpitaux et des Ehpad, une loi ambitieuse, qui place l'être humain au coeur du système de santé,

Le projet de loi que vous nous avez présenté, madame la ministre, répond-il à la détresse de ces personnes, tant dévouées et motivées et qui se mettent en arrêt maladie ? Depuis trois mois, vous n'avez pas pris la mesure d'un niveau d'épuisement rarement atteint. Ces situations humaines, tant pour les patients que pour les personnels, sont totalement insupportables. L'avenir ne se construira pas sans apporter des solutions aux difficultés du présent, ce « pressant avenir immédiat », selon l'expression du philosophe Vladimir Jankélévitch.

vives, j'y insiste, madame la ministre, quand le Gouvernement ne respecte pas le dialogue parlementaire, ne respecte pas le temps nécessaire à la concertation et à l'élaboration d'un projet de loi, non plus que le temps nécessaire pour imaginer les solutions les plus innovantes avec les acteurs de la santé et les élus. Alors que le Premier ministre s'était engagé à mieux écouter les Français, à renforcer le dialogue avec les corps intermédiaires et les élus locaux et nationaux, vous êtes déjà rattrapée par vos vieux démons.

à la procédure d'urgence, vous nous demandez de renoncer au débat parlementaire et de vous autoriser à légiférer par ordonnances. encore, affirmait pourtant, lundi 8 avril, qu'il souhaitait renforcer le dialogue avec les élus, et qu'il entendait construire « les outils d'une démocratie plus délibérative et participative ». Il ajoutait : « si on ne prend pas le temps d'écouter, généralement, on n'écoute pas bien.

effet, ne pas voir que ce texte sort renforcé et mieux armé à l'issue de la discussion au Sénat ? Comment ne pas constater le travail utile effectué par la commission des affaires sociales ?

un amendement socialiste, portant sur le troisième cycle des études de médecine générale et de certaines spécialités démontrent la capacité du Sénat à apporter des solutions pertinentes, réalistes et efficaces à l'angoisse de nos concitoyens vivant dans les zones où la présence médicale se raréfie. Voilà comment nous pouvons dépasser les clivages politiques pour soutenir ensemble l'intérêt général. Sans brader la formation, en liant professionnalisation et lutte contre les déserts médicaux, ce sont plusieurs milliers de futurs médecins qui viendront irriguer nos territoires et participeront à relever le défi de l'accès aux soins pour tous nos concitoyens. Concernant la formation des professionnels de santé, grâce à l'adoption d'un amendement socialiste, la détermination du nombre d'étudiants reçus en deuxième et troisième reçus en deuxième et troisième années de premier cycle fera primer le critère des besoins de santé du territoire sur celui de la capacité d'accueil des facultés.

l'avancée que constitue le dispositif, introduit sur l'initiative du rapporteur, garantissant l'interopérabilité des outils numériques en santé, assorti d'un calendrier opposable, gage d'amélioration de la qualité des soins et d'une meilleure coordination des parcours de santé. Enfin, nous l'avons longuement évoqué, l'adoption d'un amendement déposé par plusieurs de nos collègues a conduit à allonger de deux semaines le délai de recours à l'IVG, afin de lutter contre les inégalités subies par les femmes. La majorité sénatoriale et le Gouvernement ont malheureusement fait le choix de la procédure, constitutionnelle certes, mais brutale, de la seconde délibération.

pour les personnels de santé et, surtout, pour les usagers, les malades, en matière d'accès aux soins. Le groupe socialiste et républicain, malgré

législatif sur la santé en dix ans intervient dans un contexte toujours plus tendu sur nos territoires, qui vivent durement les inégalités d'accès aux soins et expriment des attentes très fortes à court et à moyen termes, à court et à moyen termes, mais également dans les services hospitaliers. Je veux, à ce sujet, profiter de cette tribune pour rappeler le soutien du groupe du RDSE aux professionnels médicaux et paramédicaux, qui se démènent pour maintenir un haut niveau de service et de prise en charge malgré les difficultés rencontrées au quotidien. Il n'est pas inutile de redire que ce projet de loi n'est pas un texte de financement. Comme son intitulé l'indique, il propose une réorganisation des soins, notamment ambulatoires. Il s'agit de ne pas donner de faux espoirs à ceux qui s'attendraient, dès demain matin, à une arrivée massive de médecins qui, comme avant, s'installeraient seuls, sur le modèle d'un médecin par village ou par quartier. Ne nous mentons pas, la situation que nous connaissons aujourd'hui résulte d'un manque d'anticipation des politiques de santé successives, notamment de la baisse du entre les années 1980 et 2000, ainsi que du vieillissement de la population, de l'explosion des maladies chroniques, ou encore des aspirations des jeunes professionnels, qui plébiscitent la pratique en équipe pluriprofessionnelle. Face à ces enjeux multiples, aucune mesure, aussi forte soit-elle, ne résoudra, à elle seule, la situation. Ainsi, la suppression du, que nous saluons, s'apparente davantage à une augmentation du nombre de médecins formés et ne portera ses fruits que dans dix ou Comme je le disais précédemment, ce projet de loi a pour ambition de répondre aux attentes très fortes des Français, pour qui la santé figure toujours parmi les premières préoccupations. Il en est de même pour les élus, qui expriment le souhait d'être davantage intégrés aux processus de décision en matière de santé sur leurs territoires.

Les attentes sont également fortes du côté des professionnels de santé qui, lors de la mission que j'ai menée avec mes collègues Catherine Deroche et Yves Daudigny, nous ont fait part de leur crainte d'une suradministration de la santé au détriment du soin

de la philosophie globale du texte, qui pose un cadre souple et laisse les professionnels s'organiser sans contrainte excessive. Il faudra néanmoins renforcer l'information et l'accompagnement de ces professionnels, afin de garantir l'efficience des dispositifs existants, car c'est bien grâce à eux, et à la coopération des collectivités, que les changements attendus se matérialiseront sur le terrain.

J'insiste ainsi sur certaines mesures qui tendent à apporter des réponses à court terme en redonnant du temps médical aux professionnels : la possibilité étendue de recourir à un médecin adjoint, les simplifications relatives au statut de praticien hospitalier, le renforcement de la télémédecine, qui ouvre une voie d'accès intéressante aux soins de premier recours, ou l'évolution de certaines tâches attribuées aux infirmiers, pharmaciens et sages-femmes, qui complète la création du métier d'assistant médical. D'autres dispositions porteront leurs effets à plus long terme : la réforme des études médicales, qui permettra de former plus de médecins, de diversifier les profils des étudiants et de mieux adapter le troisième cycle aux besoins des territoires, aux réalités du métier et aux aspirations des jeunes praticiens, ainsi que la gradation des hôpitaux, avec la labellisation de 500 hôpitaux de proximité. Bien que les apports successifs de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que les précisions du Gouvernement, aient levé certains doutes, des interrogations légitimes persistent quant à la préservation d'une offre hospitalière de proximité.

Par ailleurs, les diverses mesures de transformation numérique inscrivent pleinement notre système de soins dans le XXI siècle, en facilitant les échanges d'informations par la création de l'espace numérique et en généralisant le dossier médical partagé. Enfin, les mesures de coordination, au coeur même de ce projet de loi, devraient permettre une meilleure organisation des soins, grâce à une coopération accrue entre les professionnels à l'échelle d'un bassin de vie, apportant ainsi une réponse à la question aux soins. Avant d'achever mon propos, je souhaite toutefois faire part de deux regrets à l'issue de cette première lecture. Le premier concerne le recours aux ordonnances, trop souvent utilisé. Nous comprenons qu'il faut aller vite pour répondre à l'urgence, mais certains sujets auraient mérité un débat parlementaire plus approfondi. notamment, de la question sensible des autorisations des activités de soins dans les établissements hospitaliers. Mon second regret a trait à l'instauration d'une année de stage en ambulatoire et en autonomie à la fin du troisième cycle de médecine générale.

La qualité de cette formation, que beaucoup de pays nous envient, ne doit pas être une variable d'ajustement. Le texte issu des travaux du Sénat place des outils de coordination entre les mains des professionnels, permet une gradation des soins un décloisonnement entre les praticiens et entre la ville et l'hôpital, sans pour autant céder à la facilité des mesures coercitives, dont je suis convaincue de l'inefficacité. Toutefois, sans des moyens humains, financiers et d'accompagnement à la hauteur des enjeux, le risque existe que nous ne puissions pas constater sur le terrain les effets attendus. Aussi, attentive aux moyens qui seront engagés, mais désireuse de voir ces mesures mises en oeuvre, la majorité du groupe du RDSE votera en faveur de ce texte.

et de professionnels de santé s'investissent sans relâche auprès des institutions et avec de nombreux partenaires pour trouver des solutions localement. Madame la ministre, vous lanciez vous-même, dès octobre 2017, un plan d'accès aux soins comportant des mesures essentielles qui commencent à produire

De même, l'obligation d'intégration des ressources humaines dans les GHT relève d'une marche forcée inacceptable pour beaucoup de professionnels. Chacun doit pouvoir avancer à son rythme.

Il prend en compte les déterminants à l'installation : seuls 3 % des futurs médecins souhaitent un exercice libéral isolé, 45 % d'entre eux veulent un exercice regroupé et seulement 27 % se dirigent vers un exercice mixte.

68 % des étudiants de deuxième cycle ayant fait le stage d'initiation à la médecine générale déclarent que celui-ci leur a donné envie de choisir cette spécialité. Rappelons toutefois qu'entre 2010 et aujourd'hui le nombre de médecins généralistes a baissé de près de 8 %.

d'effectuer leurs stages à l'extérieur des hôpitaux publics, notamment dans les cliniques privées et dans le secteur libéral. Les amendements identiques déposés par Corinne Imbert,

rencontrer les acteurs, relever les difficultés, comprendre les enjeux liés à chaque territoire, mettre du lien entre institutions et professionnels sont autant d'actions qui mériteraient une véritable structuration.

paramédical dans les Ehpad, mais aussi dans les hôpitaux. Je me réjouis donc que le Sénat ait adopté deux amendements du groupe centriste allant dans ce sens. Le premier visait à préciser que les intercommunalités

afin de le rendre plus efficace pour répondre aux grands enjeux de notre siècle : inégalités territoriales d'accès à la santé, vieillissement de la population et recrudescence des maladies chroniques. Ce texte a fait naître de nombreuses attentes, comme nous l'avons constaté au cours du grand débat national. Il traduit certains engagements du plan Santé présenté par le Président de la République et contient un certain nombre de réformes nécessaires, dont nous saluons l'adoption par le Sénat. Le coeur du texte réside, à mon sens, dans la résorption progressive, mais indispensable, des déserts médicaux, dans lesquels vivent six millions de Français aujourd'hui.

a proposé de transformer la dernière année de troisième cycle en année de pratique ambulatoire, en affectant prioritairement les futurs médecins vers des maisons de santé situées dans des zones à faible densité médicale. Ainsi, les 3 500 étudiants en dernière année d'études de médecine générale pourront exercer en priorité, en tant que médecins adjoints, dans les territoires qui en ont le plus besoin. Nous saluons l'adoption de cette mesure, à la fois formatrice et juste,

par la grande majorité des membres de notre assemblée. Nous avons également défendu un dispositif, adopté par le Sénat, visant à sécuriser le contrat d'engagement de service public en proposant d'aligner la durée du classement en zone sous-dense sur celle de l'internat de médecine générale. à trois ans après la thèse de la durée de remplacement, associée à un dispositif de forte incitation fiscale à l'installation rapide des jeunes médecins, va également dans le sens d'une stabilisation nécessaire des communautés médicales sur l'ensemble du territoire.

En ce qui concerne la procédure de régularisation des praticiens à diplôme hors Union européenne, les Padhue, nous approuvons l'élargissement contrôlé du dispositif, tel que le Sénat l'a adopté à l'article 21. que le mécanisme d'exonération fiscale inséré à l'article 4 par la commission des affaires sociales de la Haute Assemblée ne soit pas davantage ciblé sur les installations de jeunes médecins dans les territoires sous-dotés. Nous avions proposé un sous-amendement qui allait dans ce sens, à nos yeux, d'une précision importante pour faire de cette mesure un levier d'action supplémentaire contre les déserts médicaux. Nous regrettons également que notre proposition de rétablir le droit opposable au médecin traitant Ce nouveau droit aurait offert la possibilité de saisir le conciliateur de la caisse d'assurance maladie, afin qu'un médecin traitant disponible soit proposé, de garantir le même niveau de remboursement à chaque citoyen et de lutter contre le non-recours aux soins. Enfin, nous aurions souhaité que le Sénat examine en séance l'amendement que nous avons proposé visant à étendre le droit à l'oubli,

L'association des professionnels libéraux, des hôpitaux de proximité et des établissements médico-sociaux au travers de l'engagement des communautés professionnelles territoriales de santé dans un projet territorial de santé, en présence des élus, va dans le bon sens. Il s'agira aussi, pour l'ARS, d'accompagner les acteurs de terrain, sans créer de rigidités ni de nouvelle strate administrative, pour améliorer le fonctionnement de notre système de santé et répondre aux attentes légitimes des Français. Nous devons faire des hôpitaux de proximité un pivot essentiel de l'articulation des soins à l'échelle du territoire en organisant une réponse graduée aux besoins de santé des patients

et améliorer l'accès à la santé pour tous ; considérant que le Sénat a largement contribué à en améliorer les dispositions, notamment pour mieux lutter contre les déserts médicaux, le groupe Les Indépendants-République et

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, avec près de 250 amendements émanant des différents groupes, adoptés en commission des affaires sociales puis en séance, le Sénat a contribué, dans un esprit constructif, à enrichir ce projet de loi. Je tiens à saluer en particulier le travail du rapporteur, le président Alain Milon, et des rapporteurs pour avis, Laurent Lafon et Jean-François Longeot. Par-delà nos divergences, nous avons tous eu à coeur, lors de cette semaine de débats souvent passionnés, de traduire dans ce texte l'urgence d'agir pour refonder un système de santé à bout de souffle. Cette urgence, les membres du groupe Les Républicains l'entendent dans les territoires depuis de trop nombreuses années. Les inquiétudes voire le sentiment d'abandon qu'expriment nos concitoyens sont à la mesure de leur attachement fort à notre modèle de prise en charge solidaire des soins. Au regard de ces attentes pressantes, nous avons été nombreux à formuler des regrets sur le projet de loi transmis au Parlement. Le regret, d'abord, de discuter d'un texte qui laisse un sentiment d'inachevé et bon nombre d'interrogations en suspens, puisque ce sont des ordonnances qui donneront le ton de la réforme, y compris pour des mesures essentielles. Le regret, ensuite, de ne pas trouver dans ce texte des éléments structurants sur la gouvernance ni le financement de notre système de santé, car des enjeux majeurs pour l'avenir de notre modèle de prise en charge des soins Toutefois, nous avons reconnu des inflexions positives, que nous avons cherché à améliorer et à approfondir. Le texte issu de nos débats confirme des évolutions attendues, comme la refonte des études de santé, qui permettra une sélection plus progressive des futurs professionnels médicaux et une diversification de leurs profils. Il confirme également la nécessité urgente de faire entrer notre système de santé dans l'ère numérique. Nous pouvons saluer le travail accompli par la commission des affaires sociales et, plus généralement, le Sénat pour enrichir substantiellement ce volet en rendant automatique l'ouverture de l'espace numérique de santé, tout en prenant en compte les enjeux de protection des données, de médiation numérique et, surtout, les exigences d'interopérabilité. Les enjeux sont considérables pour faciliter les transmissions d'informations et constituer un levier pour l'indispensable coordination des parcours de soins.

La réforme du limitera sans doute le gâchis universitaire de la Paces pour bon nombre d'étudiants, et c'est heureux ; mais elle ne conduira pas demain à ce qu'il y ait plus de médecins dans les cabinets médicaux et les hôpitaux. De même, la redéfinition des hôpitaux de proximité ne se fera pas sans ressources médicales, sauf à accélérer le déclassement d'établissements locaux, tant redouté par de nombreux élus. Nous savons bien qu'il n'existe pas de solution miracle pour répondre à l'urgence de la présence médicale dans les territoires. J'entends les arguments avancés par chacun sur les stages, le conventionnement sélectif ou les autres modalités de contrainte ou de régulation des installations.

nous voulons négocier avec les médecins sur leur contribution à la réduction des inégalités territoriales. Enfin, nous avons prévu de professionnaliser la dernière année d'internat de médecine sous la forme d'une pratique ambulatoire, en autonomie, qui se déroulerait en priorité dans les zones sous-dotées.

J'entends les réserves de jeunes étudiants, qui craignent que cela ne conduise à raboter leurs études et la qualité de leur formation, mais je pense, au contraire, que la professionnalisation fait partie de leur formation. Il n'appartient toutefois qu'à vous, madame la ministre, d'inscrire cette proposition dans la rénovation des études médicales, pour faire de cette année sur le terrain une réponse au besoin des jeunes praticiens d'être mieux accompagnés dans la construction de leur projet professionnel.

viendraient en renfort à court terme, au côté de médecins installés, sur les territoires fragilisés en termes démographiques, soit, en moyenne, trente-cinq médecins par département.

de l'organisation territoriale de la santé, notre conviction s'appuie sur la confiance faite aux acteurs de terrain. Nous avons été nombreux à plaider pour la souplesse et la simplification contre la tentation d'une hyperadministration de la santé. Ne décourageons pas les porteurs de projet en les enferrant dans des carcans trop rigides. Selon la même logique, nous avons privilégié les démarches de volontariat des établissements pour poursuivre l'acte II des groupements hospitaliers de territoire. Nous avons souhaité également rééquilibrer les rôles de l'État et la région, au travers des agences régionales de santé et des élus du territoire, en renforçant les prérogatives du conseil de surveillance de ces agences et en en confiant la présidence à un élu, le président de région.

Le texte qui résulte de nos travaux offre des réponses concrètes, complémentaires, simples sans être simplistes, nourries de notre vécu. Madame la ministre, écoutez la voix du Sénat, car elle exprime notre souhait à tous de voir réussir cette réforme, pour moderniser un système de santé en crise et répondre à l'urgence des territoires et à l'appel de nos concitoyens. Le groupe Les Républicains votera le projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé tel que le Sénat l'a modifié ! Très bien ! Mes chers collègues, il va être procédé, dans les conditions prévues par l'article 56 du règlement, au scrutin public solennel sur l'ensemble du projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé. Ce scrutin, qui sera ouvert dans quelques instants, aura lieu en salle des conférences, parallèlement aux explications de vote sur la proposition de loi visant à permettre aux conseillers de la métropole de Lyon de participer aux prochaines élections sénatoriales. Je remercie nos collègues Annie Guillemot, Michel Raison et Patricia Schillinger, secrétaires du Sénat, qui vont superviser ce scrutin. Je rappelle qu'une seule délégation de vote est admise par sénateur. Je déclare le scrutin ouvert pour une durée maximale de trente minutes et vais suspendre la séance pour quelques instants.

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle les explications de vote et le vote sur la proposition de loi visant à permettre aux conseillers de la métropole de Lyon de participer aux prochaines élections sénatoriales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

depuis le 1 janvier 2015, la métropole de Lyon remplace la communauté urbaine de Lyon et, dans son périmètre, le département du Rhône. Un département, le Nouveau-Rhône, subsiste néanmoins, en dehors des limites de la métropole. Contrairement aux autres métropoles, celle de Lyon est non pas un établissement public de coopération intercommunale, un EPCI, à fiscalité propre, mais une collectivité territoriale à statut particulier, régie par l'article 72 de la Constitution. Elle exerce les compétences d'un département et certaines compétences des communes. À compter de mars 2020, le conseil de la métropole de Lyon sera composé de 150 membres, élus au suffrage universel direct. est prévu pour les EPCI, la représentation des communes n'y sera plus garantie, ce qui soulève de réelles difficultés sur le terrain. La proposition de loi de François-Noël Buffet et de plusieurs de ses collègues vise un objectif plus immédiat corriger une malfaçon du code électoral pour permettre aux conseillers de la métropole de Lyon de participer aux prochaines élections sénatoriales, prévues en septembre 2020.

Le corps électoral compte 3 500 grands électeurs, dont 3 410 issus des conseils municipaux. En l'état du droit, les conseillers de la métropole de Lyon ne peuvent pas participer aux élections sénatoriales. En effet, ils ne figurent pas dans la liste des grands électeurs établie à l'article L. 280 du code électoral. Cette situation n'a pas été souhaitée par le législateur. Elle résulte d'une erreur de coordination de l'ordonnance du 19 décembre 2014, comme l'a confirmé le secrétaire d'État en commission. elle soulève un fort risque contentieux. En effet, en application de la jurisprudence constitutionnelle, l'élection des sénateurs doit respecter trois critères : l'élection par des élus locaux, la représentation de l'ensemble des collectivités territoriales et la prise en compte de la démographie. dans le Rhône, ces deux derniers critères ne sont plus respectés : la métropole de Lyon n'est pas représentée pour l'élection des sénateurs, alors qu'elle constitue une collectivité territoriale à statut particulier et compte 1,35 million d'habitants. la présente proposition de loi autorise les 150 conseillers de la métropole de Lyon à participer aux élections sénatoriales. Elle entrerait en vigueur dès le prochain scrutin, prévu en septembre 2020. Le nombre de grands électeurs dans le Rhône passerait ainsi de 3 500 à 3 650, soit une augmentation de 4,29 %. Cette proposition de loi me semble indispensable pour sécuriser les élections sénatoriales dans le Rhône. Elle comble opportunément une lacune du code électoral : en tant qu'élus locaux, les conseillers de la métropole de Lyon ont vocation à participer aux élections sénatoriales. L'enjeu est double sur le plan juridique, il s'agit de respecter la jurisprudence constitutionnelle, qui impose que toutes les catégories d'élus locaux participent aux élections sénatoriales ; sur le plan politique, il convient d'assurer une certaine équité entre les conseillers métropolitains et les autres élus locaux. Ce texte fait consensus entre les sénateurs du Rhône- je l'ai constaté lors de mes auditions. Ainsi, selon notre collègue Michel Forissier, il est indispensable pour réparer une inégalité de traitement entre élus. Je rappelle que nous devons agir rapidement : sauf modification liée aux réformes institutionnelles, les prochaines élections sénatoriales dans le Rhône auront lieu dans tout juste quinze mois. cette proposition de loi ne modifiera qu'à la marge les élections sénatoriales dans le Rhône : les 150 conseillers de la métropole de Lyon, qui seront issus de différentes familles politiques, ne représenteront que 4,11 % du collège électoral. La commission s'est interrogée sur un éventuel déséquilibre démographique entre la métropole de Lyon et le département du Nouveau-Rhône. En effet, la métropole bénéficierait d'une meilleure représentation aux élections sénatoriales que le département : un conseiller métropolitain représenterait 9 030 habitants, contre 17 208 pour un conseiller départemental. Après analyse, cette situation semble compatible avec la jurisprudence constitutionnelle, quelle que soit l'interprétation retenue. Selon une première interprétation, la métropole et le département représenteraient deux strates de collectivités distinctes, la métropole exerçant les compétences d'un département, mais également certaines compétences des communes. Dans une telle hypothèse, la jurisprudence constitutionnelle n'impose pas de prendre en compte la population respective de la métropole et du département pour répartir les grands électeurs. Selon une seconde interprétation, la métropole et le département appartiendraient à la même strate de collectivités territoriales. La jurisprudence constitutionnelle reste toutefois relativement souple : elle

la ville de Lyon, par exemple, est moins bien représentée que les communes rurales, ce qui permet de représenter plus équitablement les territoires au sein de notre assemblée.

une nouvelle collectivité territoriale à statut particulier a été créée par la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite loi Maptam : la métropole de Lyon. La nouvelle collectivité territoriale est dotée de pouvoirs importants, puisqu'elle assume sur le territoire de l'ancienne communauté urbaine de Lyon certaines compétences des communes et toutes les compétences du conseil départemental. Cet acteur majeur du territoire est aussi un acteur politique, avec pour instance de gouvernance un conseil métropolitain de 150 membres, élus au suffrage universel direct : ils seront désignés, pour la première fois, concomitamment aux élections municipales de mars prochain.

Concrètement, l'ordonnance de 2014, prise en application de la loi Maptam, n'a pas ajouté la mention des élus du conseil métropolitain de Lyon à l'article L. 280 du code électoral. L'effet de cette absence est direct : si les élections sénatoriales se tenaient demain, en l'état du droit, les conseillers métropolitains de Lyon n'auraient pas le droit de vote. Cette situation ne pouvait pas durer, avant tout parce qu'elle provoque un problème majeur de non-représentation politique.

dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales », mais aussi à la Constitution, puisque le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 6 juillet 2000, 2000, a été plus explicite encore, jugeant que le Sénat devait être élu par un corps électoral représentant toutes les catégories de collectivités territoriales.

Il me paraît atteindre simplement et efficacement l'objectif qu'il vise : inscrire les conseillers métropolitains de Lyon sur la liste des grands électeurs pour les élections sénatoriales.

Son identité n'est pas achevée, et plusieurs modèles se profilent, comme l'ont souligné mes collègues Claude Raynal et Charles Guené dans leur rapport d'information. « Affaire d'hommes

de la conférence des maires, seule instance où ces derniers siègent en tant que tels. Nous voulions renforcer aussi le pouvoir de consultation des conférences territoriales, déclinaisons locales de la conférence des maires.

l'adapter à la métropole de Lyon, grâce à un amendement de Mme Annie Guillemot. Cet après-midi, nous débattons de nouveau d'un sujet technique lié à cette institution originale. Ne serait-il pas temps de se poser la question d'un texte spécifique pour une métropole à statut spécifique ? dans le cadre d'un grand texte général, et non par une accumulation de corrections techniques ! Cela nous donnerait l'occasion de nous interroger sur les conséquences en termes de gouvernance de ce statut particulier particulier et de réfléchir ensemble à des questions aussi importantes que celle des échelons de proximité entre la métropole et ses habitants. Sans proximité, la métropole risque un destin proche de celui de l'Union européenne

Cette réflexion peut avoir lieu à l'occasion d'une future réforme de la décentralisation annoncée par le Président de la République ou plus tard, après une phase d'évaluation à l'issue du prochain mandat. Mais un texte de portée générale sur la métropole de Lyon fait

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, conjointement à la tenue des prochaines élections municipales, les électeurs du Grand Lyon seront amenés à élire, dans le cadre d'un scrutin distinct, leurs conseillers métropolitains. Depuis le 1 janvier 2015, date de la création de la nouvelle collectivité territoriale à statut particulier dénommée « métropole de Lyon », ce sont les anciens conseillers de la communauté urbaine qui siègent toujours en son sein. Ces derniers, comme tous les conseillers communautaires de France, sont susceptibles d'être parties prenantes du corps électoral aux élections sénatoriales de par leur mandat communal, ayant été désignés dans le cadre d'un fléchage. Or le prochain renouvellement des conseillers métropolitains lyonnais devant désormais se faire dans le cadre d'un scrutin supra-communal, il convient de permettre aux futurs élus d'être associés aux prochaines élections sénatoriales.

groupe du RDSE souscrit à la proposition de notre collègue Jean-Noël Buffet, laquelle répare une omission et permet une modification du collège électoral des sénateurs dans le département du Rhône. L'occasion nous est donnée de revenir brièvement sur la perspective de cette élection au sein du Grand Lyon, qui conduira, pour la première fois à l'intérieur d'une métropole, à faire exercer des compétences pour partie précédemment communales par des élus qui ne seront plus nécessairement également des élus municipaux. Le Sénat, de manière constante, a rappelé son attachement à ce que la commune demeure la cellule de base dans toute forme de coopération intercommunale. Ce lien ne saurait être rompu sans menacer la pérennité de la structure communale. Le Sénat a également pris acte du fait que, en l'état des règles institutionnelles, il n'est pas possible de garantir une représentation de l'ensemble des communes concernées au sein d'une métropole ayant acquis le statut de collectivité territoriale. Dès son élection, le Président de la République a fait part de son intention de voir reproduit le modèle lyonnais et de favoriser la fusion des compétences départementales et métropolitaines, au sein des périmètres métropolitains, dans le cadre de la création de nouvelles collectivités territoriales. Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Nice ... : plusieurs tentatives de rapprochement ont été entreprises. Elles n'ont pas pu à ce jour faire l'objet de consensus locaux, comme cela avait été le cas à Lyon. Les récents travaux de la commission des finances sur ces évolutions institutionnelles, en l'occurrence la fusion intervenue sur le territoire du Grand Lyon, ont conclu qu'une telle entreprise serait difficilement reproductible. En effet, une large part de l'équilibre du modèle lyonnais réside notamment dans le fait que la dynamique économique et financière existant autour de l'aéroport Lyon-Saint Exupéry continue de profiter au département du Rhône. Une configuration différente aurait vraisemblablement entraîné un profond déséquilibre en termes de moyens et d'attractivité. Un ultime projet de fusion demeure actif, celui de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Le Gouvernement souhaiterait le concrétiser sur l'ensemble du périmètre des Bouches-du-Rhône, écartant, notamment, ainsi le délicat sujet des ressources des territoires demeurant hors du périmètre métropolitain au sein d'un même département. Là encore, si le projet aboutit- les élus bucco-rhodaniens attendent, monsieur le secrétaire d'État, avec une impatience désormais non dissimulée les propositions du Gouvernement -, il ne sera pas possible, en l'état du droit, d'assurer la représentation de l'intégralité des communes au sein de la future collectivité territoriale. La nouvelle métropole marseillaise, comme c'est le cas à Lyon, s'emparera de compétences précédemment communales, qui affecteront largement l'action municipale. Mais toutes les communes ne pourront y être représentées ou, situation ubuesque, certaines pourraient l'être par des opposants aux maires en place. Cet écueil appelle peut-être une évolution de nos règles institutionnelles. Si l'égalité des citoyens devant le suffrage est un principe à valeur constitutionnelle, la représentation de tous les territoires doit aussi être une préoccupation du creuset qui s'installe inexorablement entre les territoires urbains, périurbains et ruraux, une diversité de territoires que l'on serait susceptible de retrouver dans la future métropole marseillaise. Au travers de la défense de l'échelon communal, le Sénat a toujours été soucieux de maintenir une véritable proximité, un lien physique avec nos concitoyens, et ce dans l'ensemble de nos territoires. Nous n'oublions pas que les Français veulent garder des élus « à portée d'engueulades » dans leurs communes, comme au Parlement d'ailleurs. La parole

de poser le sujet en rappelant certains éléments, même si les orateurs précédents les ont évoqués. En devenant le 1 janvier 2015 la première métropole à statut particulier de France et non plus un EPCI, la métropole de Lyon intégrait sur les cinquante-neuf communes de son territoire toutes les compétences du conseil départemental, tandis que le conseil départemental du Nouveau-Rhône voyait le jour pour le reste du département. Le Rhône se divise désormais en deux entités administratives distinctes : la métropole et le conseil départemental. De fait, les conseillers communautaires fléchés lors des élections municipales de 2014 ont obtenu, dans la nuit du 31 décembre 2014 au 1 janvier 2015, la double casquette de conseillers métropolitains et de conseillers départementaux. En 2020, le mode de scrutin changera, comme cela a été évoqué : le fléchage disparaîtra au profit d'une élection métropolitaine au suffrage universel direct dissociée des élections municipales, même si le scrutin aura lieu le même jour, ce qui ne sera pas sans troubler les électeurs. Les citoyens éliront donc les maires des 59 communes et les 150 conseillers métropolitains répartis sur 14 nouvelles « circonscriptions Maptam » : celles-ci sont différentes des circonscriptions législatives ; elles sont liées au poids démographique, sans tenir compte des entités communales. Il est entendu qu'il n'y a pas nécessairement de lien entre les listes : aucune obligation, par exemple, pour un conseiller métropolitain d'être présent sur une liste municipale. Dans le cadre de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, il convient d'ajuster le droit à notre spécificité, à savoir de faire des 150 conseillers métropolitains des grands électeurs lors des prochaines élections sénatoriales. Nous partageons tous, me semble-t-il, l'idée de ce nécessaire ajustement, et l'ensemble du groupe centriste votera en Permettez-moi, toutefois, de profiter de cette tribune pour remettre en perspective le volet démocratique de ce nouveau mode de scrutin, volet qu'il nous faudra corriger. J'aurais aimé le faire pour l'échéance de 2020, mais des événements malencontreux ne l'ont pas permis. je persévère pour 2026. Très simplement, il faut considérer que toutes les communes ne seront plus représentées au sein du conseil de la métropole. Pis encore, comme cela a été relevé, il est possible qu'un maire démocratiquement élu voie son opposant élections municipales, mais gagné aux élections métropolitaines siéger au conseil métropolitain et représenter sa commune. Avouons-le, cette situation sera assez incompréhensible pour les citoyens. Certains disent qu'il en est de même pour les élections départementales, à la nuance près que, dans notre cadre, les communes délèguent des compétences à la métropole comme un EPCI. Il est donc impossible de fait d'être le premier échelon de proximité sans siéger dans les organes délibérants. La contrainte juridique est actuellement liée à la logique démographique et au fameux tunnel des plus ou moins 20 %. C'est ce point qu'il conviendra de modifier et qui pourrait être étudié lors de la prochaine révision constitutionnelle. Je vous donne donc rendez-vous, mes chers collègues, et j'espère que ce texte

janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, la métropole de Lyon est une collectivité à statut particulier, qui exerce les compétences de l'ancienne communauté urbaine de Lyon, celles du département et certaines compétences des communes depuis le 1 janvier 2015. Toutefois, l'ordonnance relative à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon n'a pas prévu que les 150 conseillers qui seront élus au suffrage universel direct à compter de 2020 participent aux élections sénatoriales. Or cette situation n'a pas été souhaitée par le législateur, qui n'a jamais exprimé sa volonté d'exclure les conseillers métropolitains du corps électoral des élections sénatoriales. C'est pour remédier à cette erreur de coordination de l'ordonnance que la proposition de loi de notre collègue François-Noël Buffet autorise les 150 conseillers de la métropole de Lyon à participer aux élections sénatoriales dès le prochain renouvellement du Sénat, en 2020. Ainsi, après ajout des conseillers métropolitains, le nombre de grands électeurs dans le Rhône passerait de 3 500 à 3 650 personnes, soit une augmentation de 4,29 %- le nombre exact n'est pas connu à ce jour, car il faut attendre le dernier le dernier relevé de l'Insee. Cette proposition de loi paraît pertinente, puisqu'elle vise à sécuriser les élections sénatoriales en levant un risque contentieux. Elle répond à un double enjeu. En premier lieu, elle assure une certaine équité entre les conseillers métropolitains et les autres élus. En second lieu, elle respecte la jurisprudence constitutionnelle, qui exige que toutes les catégories d'élus locaux participent aux élections sénatoriales. Je tiens à saluer, pour la qualité de ses travaux, la rapporteure, notre collègue Claudine Thomas, qui s'est interrogée sur un éventuel déséquilibre démographique entre la métropole de Lyon, d'une part, et le département du Nouveau-Rhône, d'autre part. Aux élections sénatoriales, un conseiller métropolitain représenterait 9 030 habitants, contre 17 208 habitants pour un conseiller départemental. La rapporteure nous a rassurés sur ce point, cette situation serait compatible avec la jurisprudence constitutionnelle. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, cette proposition de loi remédie opportunément à une lacune du code électoral et fait consensus entre les sénateurs du Rhône. Le groupe Les Indépendants la votera sans réserve.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je préfère mettre fin au suspense tout de suite : nous voterons ce texte.

Si le Conseil constitutionnel n'est jamais revenu sur ce sujet, c'est parce qu'il n'aurait pas été satisfait d'avoir à juger

démographique des différentes catégories d'élus, et c'est en effet tout à fait conforme aux principes énoncés par la jurisprudence constitutionnelle. Nous n'avons donc que des raisons de nous réjouir du dépôt de ce texte, auquel nous